est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire qui sera chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique en cours d'examen.

L'organisme de logement social doit pouvoir rester libre de définir sa stratégie patrimoniale, afin de contribuer à la poursuite de l'objectif de 25 % de logements sociaux fixé par la loi SRU. En zone tendue, compte tenu de la rareté des opportunités foncières, la vente de logements sociaux ne pourra pas être compensée par la création d'autres logements sociaux. L'incitation à la vente aurait donc pour effet de freiner la progression vers l'objectif, mais aussi potentiellement, à échéance du décompte SRU fixé à dix ans, de réduire la part de logements sociaux dans la commune. Faut-il rappeler que les zones tendues manquent cruellement de logements abordables adaptés aux ressources et aux besoins des Français ? Cet amendement vise à rendre facultative la liste de logements annexée à la convention d'utilité sociale,

prévoit l'introduction d'un plan de mise en vente au sein des CUS, sachant que la signature de ces conventions vaut autorisation globale de mise en vente. Je précise que la vente au fil de l'eau est toujours possible pour des immeubles qui n'auraient pas été identifiés dans la CUS. Cette rédaction du projet de loi ne rend pas obligatoire l'inscription de logements aliénés dans le plan de mise en vente. Sur un plan juridique, Mme la rapporteur vient de le rappeler, l'organisme y expliquera son souhait de ne vendre aucun logement le cas échéant,

et de performance énergétique liée au logement mentionnée à l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation ne paraît plus suffisante. Le plan de mise en vente valant autorisation de vendre pendant six ans, sans autre encadrement ultérieur, il est proposé que les informations relatives au bâti soient renforcées au stade de la CUS. L'accession sociale à la propriété doit se réaliser dans les meilleures conditions financières, sociales et patrimoniales ; nous le voulons tous. La vente des logements ne doit ni mettre en danger la situation financière des ménages ou la qualité du bâti vendu, ni engendrer des copropriétés dégradées. cet amendement, il est proposé que le plan de mise en vente comporte, pour chaque immeuble destiné à la vente, un état descriptif de l'état du bâti et des équipements mentionnant, le cas échéant, les gros travaux réalisés au cours des cinq dernières années et les travaux d'amélioration que l'organisme prévoit d'engager avant la mise en vente des logements. Quel

le plan de mise en vente s'accompagne d'ores et déjà des documents relatifs aux normes d'habitabilité et de performance énergétique. De plus, l'état du patrimoine- c'est la situation actuelle

ou dans les autres parties de la CUS. Je ne vois pas quel serait l'intérêt d'ajouter une nouvelle disposition législative pour redire la même chose.

Le projet de loi prévoit que le plan de mise en vente comprend la liste des logements, par commune et par EPCI, que l'organisme de logement social prévoit d'aliéner pour la durée de la convention d'utilité sociale, ou CUS. Ce plan de vente valant autorisation de vendre pendant la durée de la CUS, l'organisme est tenu de consulter la commune d'implantation et les collectivités qui ont accordé un financement ou leur garantie d'emprunt. La consultation de la commune d'implantation nous paraît évidemment essentielle : c'est la commune qui impulse la construction de logement social sur son territoire, et c'est à elle de décider de sa politique de logements sociaux. Les collectivités qui ont accordé des financements et leur garantie d'emprunt sont également consultées, mais l'accord de ces collectivités est essentiel à ce stade puisque, en tout état de cause, elles devront donner leur accord au transfert de la garantie d'emprunt. Il est donc proposé de préciser que la consultation concerne les collectivités et leurs groupements, afin de viser expressément les EPCI qui accordent leur appui aux opérations de réalisation de logement social et qui pilotent le PLH.

de s'opposer à la vente des logements sociaux sur sa commune. Si nous insistons sur l'importance de mettre en place cet avis conforme

supprimer l'avis conforme du maire et des EPCI sur la vente de logements, en rappelant qu'il s'agit de l'état actuel du droit et qu'il n'y a pas lieu de changer les règles. C'est oublier, monsieur le ministre, les objectifs de ventes de logements sociaux, voire d'immeubles entiers. Les logements seront vendus à leurs locataires, mais également à des sociétés de vente d'HLM, et même à des sociétés privées. Ce changement de cap va avoir des effets importants sur l'activité des organismes d'HLM et la politique du logement dans les territoires. La commission a adopté à la quasi-unanimité une mesure sur la nécessité de requérir l'accord du maire et des EPCI avant toute vente massive de logements sociaux dans leur territoire, ce qui nous semble de bonne gestion.

vous supprimez la taxe d'habitation, c'est-à-dire le lien entre les habitants et la mairie. Tout à fait ! Désormais, très logiquement,

étaient parfaites, s'il n'existait strictement aucun problème dans le domaine du logement, de la construction de logements sociaux dans ce pays, ça se saurait

l'un des consensus consistait à dire qu'il fallait redonner le pouvoir aux maires, car les maires se sentent dépossédés de ce qui fait l'essence de leur condition et de leur pouvoir dans une commune, c'est-à-dire le droit de l'urbanisme.

cet avis conforme, même si, comme mes collègues l'ont dit, on n'était pas dans le même contexte, avec le même nombre de ventes de logements sociaux. Ensuite, je voudrais dire que je comprends parfaitement votre position, monsieur le ministre : vous ne souhaitez pas que les maires

monsieur le ministre.

dans mes intentions de fragiliser ou de remettre en cause le pouvoir des maires en matière de permis de construire.

à la suite de plusieurs amendements identiques, et notamment- je tiens à le souligner -d'un amendement de la commission de la culture, a considéré que rien ne justifiait d'exclure totalement les bailleurs sociaux

Ses promoteurs pensent ainsi que s'exonérer des concours d'architecture, c'est gagner du temps et de l'argent. Rien n'est moins sûr, en réalité. Cet article est une illustration très simple de cette volonté de déréglementation et de dérégulation de l'urbanisme et de la construction. Tout irait tellement plus vite si les promoteurs pouvaient délivrer eux-mêmes les autorisations d'urbanisme, pratiquer les révisions des plans locaux, faire des plans de construction, diriger la construction, les travaux, gérer les locataires, et j'en passe ! Tout cela n'est pas sérieux, mes chers collègues. La responsabilité publique est importante, surtout lorsqu'il s'agit de l'accès au logement. Si le concours d'architecture a été instauré, c'est parce qu'il répond à un enjeu d'utilité publique. Les normes ont historiquement permis de faire des progrès importants en matière de sécurité, de salubrité, de confort et de performance énergétique.

Or, ceux-ci étant habitués à des logiques de commercialisation classique, leur production tend à une uniformité de forme architecturale qui appauvrit les villes. Ils sont plus intéressés par la rentabilité de l'opération que par sa pérennité, contrairement aux architectes. Dans ce processus, l'architecte ne tient souvent d'exécutant qui se limite à optimiser le rendement de plan et à rechercher les solutions les plus économiques, souvent en partie au détriment de la qualité. Le risque, avec la disparition du concours, est que les bailleurs sociaux finissent par s'aligner sur la manière de faire des promoteurs et perdent ce qui fut un de leur grand mérite au cours du siècle passé : être les fers de lance de l'architecture, de l'innovation et du progrès.

Pourtant, cette assertion ne résiste pas à une étude objective et poussée. Depuis la réforme de la commande publique de 2016, il est observé que le délai moyen entre la publication de l'avis initial et la désignation du lauréat est de 225 jours. À titre comparatif, les procédures négociées nécessitent environ 230 jours et, pour la conception-réalisation dont nous avons parlé hier, le délai est porté à 350 jours. jours. Il est important également de souligner que le concours permet aux bailleurs de disposer, dès la signature du marché, d'études de conception ou d'un avant-projet sommaire- le fameux APS -qui raccourcissent les délais et facilitent l'enchaînement rapide vers le dépôt du permis de construire, à l'inverse des autres procédures.

l'indemnisation des groupements non retenus représente environ 1,4 % du montant du marché et la somme des primes en concours constitue, en moyenne, 0,68 % de l'enveloppe financière réservée aux travaux par les bailleurs. Par conséquent, rapporté au coût d'une opération, le montant apparaît vraiment assez infime.

qui semble nécessaire pour que les bailleurs sociaux restent exemplaires et pour construire des logements de qualité. D'abord, le concours participe à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions.

pour des raisons uniquement économiques, se limiter à une uniformisation de réalisation- rien de pire que des blocs qui se ressemblent et se succèdent Les détracteurs du concours d'architecture pensent que cela allonge les délais d'opération et coûte cher. Or, en général, la moyenne entre l'étude de terrain et la livraison de logements est de cinq ans.

compris entre six et huit mois pour la réalisation des projets de construction de logements sociaux. Elle limite

nettement supérieure ne serait-ce qu'à celle des opérations des promoteurs privés. Pour toutes ces raisons, nous avons considéré que les concours d'architecture pouvaient être supprimés. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent plus du tout

Monsieur Sueur, nous n'avons pas changé, ni l'un ni l'autre ; vos interpellations sont habituelles et mes réponses à vos interpellations

d'architecte. Comme l'a justement rappelé Mme la rapporteur, entre 2010 et 2016, il n'a pas été démontré que la qualité architecturale s'est effondrée dans ce pays, bien au contraire d'ailleurs,

Les mesures visant à renforcer la maîtrise d'ouvrage social pour maintenir la production ont engendré de vives réactions émanant de l'ordre des architectes. Il nous paraît essentiel de mettre fin à ces contrevérités. L'assouplissement des règles est présenté à tort comme un risque en matière de qualité architecturale et de transparence de la maîtrise d'ouvrage. Or il n'en est rien. » Ce n'est qu'une opinion, certes,

pas s'abriter chaque fois derrière l'exemple de la qualité architecturale que l'on mettrait en danger. Arguer

Je n'ai jamais entendu autant de déclarations contre l'architecture, contre l'architecture, contre cette liberté essentielle, ce droit à la création dont a parlé éloquemment Mme Sylvie Robert. Je tiens à dire les choses comme elles sont, madame le rapporteur, même si cela ne vous plaît pas. J'ai présidé de nombreux concours d'architecture. Je l'ai toujours fait avec passion et équité,

aucun argument véritable. Madame le rapporteur, on pourrait de surcroît tout à fait réformer ces concours. On pourrait décider, pour les logements sociaux, d'organiser des concours nationaux avec de jeunes architectes, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette prime à des architectes notoires

Et ce ne sont pas les brouhahas qui vont m'intimider ! Je suis sénatrice de France, mais je suis aussi sénatrice de Martinique. J'ai été élue par des élus martiniquais dans un pays particulier qui s'appelle la Martinique, qui compte moins de 370 000 habitants qui souffre de dépeuplement chronique- 3 000 à 4 000 personnes par an ! Les élus que nous sommes nous battons tous pour inverser cette tendance mortifère d'un pays qui, à terme, risque de ne plus exister.

N'oublions pas que l'urbanisme et l'aménagement doivent être inscrits dans le durable. Ce ne sont que des oeuvres que nous transmettons aux générations qui vont nous suivre. Oui au concours d'architecture

auquel j'appartiens considère que le maintien du concours est la garantie absolue de qualité. Par discipline, je voterai comme mes collègues, une fois n'est pas coutume. Mais je veux défendre le point de vue de l'USH, que vous avez lu, monsieur le ministre.

part, les discours du week-end, les professions de foi des candidats aux élections et les nombreux articles consacrés à la dictature des normes et des règlements et, d'autre part, les travaux pratiques du lundi au vendredi, où les obligations diverses et les contraintes multiples sont soutenues au détriment de la confiance que nous devrions accorder aux responsables locaux, lesquels font vivre nos territoires, qu'il s'agisse des élus ou des socioprofessionnels. En conséquence, je voterai contre des amendements par lesquels on veut par trop corseter les responsables locaux et décider ce qui est bon pour eux

Il s'agit ici d'introduire la vente dans le champ des opérations couvertes par la concertation. En l'état actuel, les opérations de construction-démolition, ainsi que celles de réhabilitation font l'objet d'une procédure spécifique spécifique : réunions publiques d'information avec les locataires et concertations avec les associations représentatives des locataires. À l'heure de la démocratie participative, il est important que les locataires et leurs représentants soient associés, par une concertation, à la mise en vente de leur immeuble,

en posant dans le code de la construction et de l'habitation le principe d'une évolution des loyers prenant en compte l'évolution de l'IRL, l'indice de référence des loyers. Le présent amendement ouvre la faculté pour les organismes d'HLM d'appliquer le loyer révisé en masse et pas seulement en valeur en ce cas, la hausse globale des loyers pratiqués de l'organisme pour l'année à venir ne peut dépasser, en masse, la variation de l'IRL. Cette disposition permettra de moduler le niveau des loyers afin de s'adapter au mieux à la réalité locale des logements et à la situation des locataires. Quel est l'avis de la commission ? au détriment du parc privé, sans que cela se justifie véritablement. Il résulte de cet amendement une rupture d'égalité entre les locataires des différents parcs. De plus, si, pour un même bailleur social, certains loyers subissent une hausse supérieure à l'IRL, d'autres

car il est aujourd'hui nécessaire que les locataires et leurs représentants soient davantage associés aux décisions qui concernent leur habitat. Dans cet objectif, le présent amendement actionne deux volets. Le premier vise à harmoniser les conditions de représentation des locataires dans l'ensemble des organismes d'HLM. d'HLM. Le second vise à porter à un tiers le nombre et la proportion des représentants des locataires siégeant dans les conseils d'administration ou de surveillance des organismes d'HLM, ainsi que dans les conseils d'administration des offices publics de l'habitat et des sociétés d'économie mixte. Les locataires sont les premiers concernés

deux observations fondamentales. Sur le fond, il est nécessaire de revoir le fonctionnement, le règlement intérieur, les conditions dans lesquelles les dossiers sont instruits et les décisions, prises.

du monde des bailleurs et des collectivités, pour simplifier et accélérer les procédures de rénovation urbaine. C'est plus qu'une déclaration d'intention, puisque, au conseil d'administration du 25 mai, déjà, un certain nombre de modifications ont été décidées et immédiatement mises en application. J'entendais, depuis que je suis en charge, avec le secrétaire d'État, de cette responsabilité, une immense majorité de représentants de collectivités locales se plaindre : « ce n'est plus possible » ; « cela dure trop longtemps » ; « on passe de véritables examens où l'on juge nos propositions, où l'on nous renvoie » en fait de système partenarial, c'est le préfet qui part à Paris plancher, alors que la collectivité reste sur place le tout avait abouti au fait que, ces dernières années, le système n'était pas totalement bloqué, mais il était grandement freiné. C'est, je crois, une constatation générale. Des décisions ont été prises, qui ont permis de simplifier

reste un problème de gouvernance. Aujourd'hui, il y a une gouvernance avec 36 membres, si ma mémoire est bonne, dont 18 représentants de l'État. Il subsiste un problème

profondément le processus, dont d'aucuns, qui ont une longue expérience de la politique de la ville, avaient dit publiquement qu'il était bloqué.

madame Létard, pour explication de vote. vos explications et votre volonté de converger vers quelque chose de plus équilibré. J'ai bien entendu également le message sur une volonté d'aboutir en CMP, mais, comme notre rapporteur m'encourage à le faire, je vais maintenir l'amendement, tout simplement pour que l'on ait une base de discussion en CMP

un certain nombre d'acteurs qui auraient toute légitimité à s'exprimer de façon équitable entre les trois collèges. Il faut un juste milieu. S'agissant des sites d'intérêt régional, veillez quand même à ce que l'argent de l'État

les ordonnances sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires et tout ce qui peut être intégré dans une agence beaucoup plus vaste. Tout cela doit se faire dans un dialogue entre

». On risque d'aboutir à une sous-représentation des collectivités locale. Par ailleurs, je pense que l'État, dans sa fonction de garant de la cohésion nationale,

comme l'ont souligné Annie Guillemot et Valérie Létard dans leur rapport sur l'application de la loi de programmation de la politique de la ville, le nouveau programme national de renouvellement urbain connaît quelques difficultés de mise en oeuvre, c'est le moins que l'on puisse dire. Afin d'y remédier, le présent amendement vise vise à faciliter le fonctionnement de l'ANRU en la soumettant à une comptabilité privée, et en adaptant certaines modalités spécifiques d'organisation et de contrôle économique et financier de l'agence. Quel est l'avis du Gouvernement ? L'avis est

globale de l'État, car, vous l'avez très bien dit, monsieur le ministre Daubresse, s'il y a eu ces accumulations de contraintes administratives, c'était pour freiner

entre les professionnels du droit et leurs clients pour des prestations soumises à tarif réglementé. C'est tout à fait le bon véhicule. Aussi, je m'engage, si Mme la présidente Primas en est d'accord, à ce que la commission des lois et la commission des affaires économiques fassent une proposition sur ce sujet à l'article 11 de ce

et j'attendrai avec impatience le travail de la commission des lois. L'amendement n° 678 rectifié est retiré. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour un rappel au règlement.

très tardivement cet après-midi. Je rappelle que nos collègues députés sont censés légiférer sur le projet de loi de révision constitutionnelle. L'affaire Benalla

». Il me semblerait donc honorable que le Sénat, par la voix de son président, Gérard Larcher, exige aussi que le Premier ministre vienne s'expliquer, s'exprimer devant notre assemblée. Bien sûr, notre commission des lois s'est saisie des prérogatives d'une commission d'enquête et va entamer un travail, et nul doute que ce travail sera

ce projet de loi très important, qui mérite toute notre attention. Or le premier questeur de l'Assemblée nationale, Florent Bachelier, ce matin, sur l'antenne de Public Sénat, a déclaré que les sénateurs étaient déconnectés des territoires,

ou quand un OPH souhaitera se faire absorber par une ESH ou par une coop. Je comprends encore moins la précision selon laquelle le silence pendant quatre mois

Ainsi, le présent article prévoit la création d'un nouveau type d'organisme d'HLM : la société de vente d'habitations à loyer modéré. Le fonctionnement de ce futur outil de vente reste, malgré les efforts de la commission, assez obscur et ses missions insuffisamment définies. Par ailleurs, les bénéficiaires de ces ventes ont été élargis. Alors que le premier objectif de la vente du parc social a longtemps été la vente aux locataires, dans une volonté de favoriser les parcours résidentiels et l'accession sociale à la propriété, le présent article dénature totalement ce dispositif. Ainsi, le parc le plus attractif qu'est le PLS, s'il est construit depuis plus de quinze ans, pourra être acquis par lot par toute personne morale, donc par un promoteur.

D'ailleurs, nous notons que le nombre d'autorisations de construction de logements sociaux s'est écroulé cette année. Voici donc le deuxième étage de la fusée du dépérissement du parc social public, lancée pour laisser place au marché.

une attaque violente, qui va nous conduire à une réduction du parc social et à son appauvrissement. C'est une vision du logement social réduit à une aide aux plus démunis, alors que la force du modèle HLM en France est d'être un système ouvert qui propose une vision généraliste du logement social Avec la vente de ce patrimoine, vous préparez les copropriétés dégradées de demain. C'est à nos yeux une politique irresponsable de votre part.

que la vente de 40 000 logements sociaux par an permettra la construction de 100 000 à 120 000 logements sociaux. Ce ratio- un logement vendu pour trois construits -, qui sonne, au passage, comme une belle campagne de publicité, a été repris de nombreuses fois pour justifier la vente de notre parc de logements sociaux. J'ai donc recherché les sources de cet argument.

En guise de source est cité le rapport d'information de 2013 des députés Christophe Caresche et Michel Piron, qui lui-même cite l'audition du 22 mai 2013 sur les aides à la construction de logements sociaux. Le même argument y est soutenu par le fait que la vente de 1 % du parc social, soit 40 000 logements, dégagerait quelque 2 milliards d'euros, permettant la construction de trois fois plus de logements neufs. Or il se trouve que c'est exactement la phrase qu'a prononcée Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme la présidence de M. Sarkozy, qui cherchait ainsi à justifier les accords de 2007 qui fixaient un objectif identique à celui d'aujourd'hui, de 40 000 ventes par an. En plus de reprendre cet objectif, fondé à l'époque sur le nombre d'HLM restant à vendre au 31 décembre 2007, le Gouvernement reprend donc le même argument lorsqu'on se penche sur cet argument vieux de onze ans et utilisé aujourd'hui pour justifier cet article 29, on s'aperçoit qu'il n'est issu ni d'une étude scientifique ni de statistiques sérieuses, mais d'une prévision très hypothétique. Celle-ci reposait sur trois prérequis que lesdites ventes génèrent 2 milliards d'euros- cela représente tout de même 50 000 euros de plus-value nette par logement -, que ces 2 milliards d'euros permettent l'octroi de 8 milliards d'euros de prêts à la construction par les banques, et surtout que la totalité de la plus-value effectuée par les sociétés de vente d'HLM soit réinvestie dans la construction. Si l'on peut fortement douter que de tels prérequis soient satisfaits dans le futur- ils ne l'ont d'ailleurs pas été à l'époque -, ils sont surtout issus d'une autre décennie et totalement obsolètes : ni le marché du logement social ni les conditions d'octroi de prêts par les banques ne sont identiques à ceux de 2007.

Je dois avouer que tous ceux qui, parmi nous, sont ou ont été élus locaux restent pantois devant une telle décision. L'évaluation des domaines sert de référence ; c'est un cadre et une garantie de transparence pour les locataires accédant

Cette logique spéculative risque d'appauvrir rapidement les plus fragiles et de menacer dans ses fondements le droit au logement. Notre amendement est simple il s'agit de rétablir l'avis des domaines dans le cadre de la vente des logements à leurs occupants. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

Le portage financier envisagé pour la vente de logements sociaux n'apporte aucune garantie pour une accession sécurisée à la propriété par les ménages les plus modestes. Il ne garantit pas non plus la bonne gestion et la pérennité du patrimoine concerné.

Qui se soucie de l'avenir de ces futures copropriétés et du sort de leurs habitants ? Les politiques de vente massive du parc social menées ces dernières années en Europe n'ont eu pour effet que de dégrader la situation du logement social, notamment dans les métropoles. D'autres solutions, en particulier au sein des regroupements qui sont mis en place, auraient pu être recherchées. Elles auraient permis d'éviter des montages qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et vont irrémédiablement affaiblir le logement social en France. Au travers de cet amendement, nous proposons donc de supprimer la création des sociétés de vente d'HLM.

et la société de vente d'HLM à se mettre d'accord sur l'entité qui prendra à sa charge les différents travaux qui devraient être éventuellement réalisés dans les logements vendus.

comme le prévoit cet amendement ; nous avons préféré apporter des précisions quant à leur fonctionnement. Je rappelle aussi que le recours à ces sociétés ne sera pas obligatoire : les organismes

s'agit d'éviter que le recours à une société de vente n'ait pour conséquence un sous-investissement sur le patrimoine avant la revente, et surtout en l'absence de revente rapide. la société de vente devra déléguer la gestion du patrimoine acquis à un bailleur social ou à un syndic, et que le contrat entre la société de vente et son et son prestataire devra préciser les modalités de prise en charge et d'exécution des travaux nécessaires pour que le programme prévu par la société de vente soit effectivement mis en oeuvre et exécuté, au besoin sous la surveillance du gestionnaire.

C'est leur patrimoine. Ce sont les Français qui ont financé la construction du logement social ; autoriser la vente de ce qui a été financé par nos compatriotes à des

de générer rapidement des fonds. L'objectif est bien de compenser la baisse des ressources qui a été imposée aux organismes d'HLM et qui menace à très court terme l'équilibre économique des organismes. Compte tenu de l'urgence, le Gouvernement autorise la cession en bloc de logements sociaux aux sociétés de vente d'HLM, mais également à des sociétés privées.

pour notre part que tous les logements sociaux, quel que soit leur financement, doivent rester dans le parc HLM. Notre amendement vise donc à prévoir que la vente en bloc ne peut se faire qu'au profit d'un organisme de logement social, et jamais au profit d'un investisseur privé.

vise à permettre aux bailleurs sociaux de valoriser plus facilement leur patrimoine. Elle conduira par ailleurs à l'instauration progressive d'une plus grande mixité sociale dans les bâtiments concernés. J'ajoute que la vente en bloc est une condition essentielle du dispositif, car

Cette mesure va à l'encontre des objectifs de réalisation de logements sociaux prévus au titre de la loi SRU. Il convient donc de faire en sorte que les ventes en bloc ne puissent pas être mises en oeuvre dans les communes carencées en logements sociaux. Il s'agit en quelque sorte d'un dispositif de protection par l'élaboration d'un cadre plus restreignant.

un PLH, du réinvestissement par l'organisme de logement social du produit de la vente d'HLM sur le territoire des collectivités concernées par un projet de vente. Ce réinvestissement se fait en faveur des politiques du logement, conformément au PLH. Il semble en effet logique que les collectivités ayant contribué au financement de la production des logements sociaux, plus globalement au financement des politiques de l'habitat, puissent bénéficier

à obtenir 30 % de logements sociaux, ce n'est pas en dix ans qu'elles pourront récupérer la perte des logements qui auront été mis en vente et qui ne seront plus comptabilisés. L'amendement n° 1014 rectifié, présenté

ne garantit en rien que les sommes issues de la vente des logements HLM soient réinvesties dans la construction de logements sur la même commune. C'est encore plus vrai dans les territoires carencés ou dans les territoires sous tension. concernées sont souvent celles qui ont les logements sociaux les plus attractifs avec un prix au mètre carré très élevé, logements susceptibles par conséquent d'être vendus très facilement. Ce sont aussi les communes où il est plus difficile de construire de nouveaux logements sociaux, par manque de foncier

On touche à la loi SRU, si l'on prend le risque d'une diminution nette de logements sociaux dans les territoires qui en ont déjà peu. Il est important de mettre en place

alors que l'offre de logement est déjà non conforme aux besoins dans ces communes qui ne semblent pas produire d'efforts pour remédier à la situation, il semble inopportun de permettre que soit encore abaissée l'offre de logements sociaux sur ces territoires. Poser un principe intelligible participe à une meilleure compréhension de la loi.

L'accession sociale répond à un souhait de nos compatriotes, mais il importe aussi que les sommes perçues soient réinvesties dans le logement social : comment s'assurer que c'est le cas, sur un même territoire ?

Compte tenu de la réorganisation des bailleurs sociaux fusionnés ou adossés à de grands groupes, il est proposé de maintenir des équilibres entre territoires tendus et territoires plus ruraux. Il est en effet nécessaire que les zones moins tendues conservent un potentiel minimal pour lancer des programmes locaux de construction et de réhabilitation. Par ailleurs, la vente des logements ne doit pas se faire au détriment des communes qui mènent depuis plusieurs années une politique ambitieuse de construction de logements sociaux. Il s'agit donc de préciser que les fonds issus des ventes de logements sociaux sont réinvestis localement,

au moins 50 % ». Ce pourcentage sera ainsi fléché vers la commune déficitaire en logements sociaux, et, lorsque la commune n'est pas déficitaire, vers la commune et l'EPCI.

de l'aliénation des logements dans les communes carencées soit affecté à la réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune carencée concernée dans un délai de cinq ans suivant l'aliénation,

Lavarde, pour explication de vote.

n'est pas vrai !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

aux conditions de cession de logements locatifs sociaux. En l'état actuel, il consacre le droit de priorité des locataires occupants au moment de l'opération,

Les sociétés de vente d'HLM définies à l'article 28 ont, entre autres, pour vocation de permettre de dégager des dividendes afin de mieux contourner la législation, laquelle tend globalement, sinon à les interdire, en tout cas à les limiter.

Dans ce contexte, le droit de préemption dévolu aux collectivités locales, singulièrement aux communes, pour les opérations de vente de logements locatifs sociaux, est le complément naturel de la législation actuelle. Je rappelle que la législation prévoit qu'une cession ne « doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive

Les nouveaux propriétaires seront des ménages par définition éligibles au logement social, ayant donc des revenus modestes. Ces personnes n'auront ainsi pas nécessairement les moyens de faire face aux coûts de rénovation de leur logement ou d'entretien de l'immeuble dans lequel est situé leur appartement.

revente. Selon nous, l'organisme vendeur doit rester pleinement engagé dans la gestion des logements, le suivi social des locataires et l'entretien de l'immeuble. Il revient à l'organisme acquéreur d'assurer les gros travaux qui incombent au propriétaire,

qu'une convention de gestion soit annexée à l'acte de vente entre les organismes HLM. Celle-ci aurait pour objet non seulement la répartition des obligations d'entretien et de travaux entre l'organisme vendeur et l'acquéreur, les modalités d'organisation des fonctions de syndic, mais également les mesures d'accompagnement mises en place pour sécuriser la vente des logements aux locataires. Quel est l'avis de la commission ?

vendre des biens publics acquis et construits avec l'argent de nos concitoyens, pour le plus grand profit du secteur privé. Nous pensons particulièrement à la future vente d'Aéroports de Paris ou à l'ancienne vente de l'aéroport de Toulouse, mais il y en a bien d'autres. La vente de logements sociaux à des particuliers eux-mêmes locataires dans le parc social pourrait s'entendre comme une politique d'aide à l'accession, l'idée de rendre possible la vente à des entreprises privées, que ce soient des banques, des assurances ou des fonds divers, apparaît comme une pure mesure opportuniste, qui offrira une rente locative à des entreprises qui n'en ont pas besoin. D'autant que seuls les meilleurs logements seront l'objet de ces achats. J'entends par là la possibilité donnée par le projet de loi de vendre des logements sociaux PLS, c'est-à-dire les plus récents, car un bâtiment construit depuis plus de quinze ans reste du patrimoine récent, et les mieux situés, les plus intéressants pour la promotion privée. On touche ici à une problématique majeure du logement social dans notre pays : même si, parmi les demandeurs, près de 75 % relèvent des plafonds de ressources correspondant

Pour résoudre ce problème d'inadéquation du parc social, du fait des ressources des demandeurs et de la construction de logements PLS plutôt que de logements PLAI, nous aurions préféré non que la vente de logement PLS soit encouragée, mais plutôt que ces logements fassent l'objet d'un reconventionnement, afin de les rendre abordables à la majorité des demandeurs de logements sociaux. Les investisseurs institutionnels devraient,

fait de permettre la vente de logements PLS, sans réels garde-fous, à des entreprises de droit privé donne libre cours à la possible spéculation, d'autant que ces logements, souvent mieux situés, peuvent susciter un réel attrait.

alinéas ouvrent la possibilité à toute personne physique d'acheter les logements vacants commercialisés par les organismes d'habitations à loyer modéré. À l'opposé de cette vision libérale, notre amendement vise à faire de la vente HLM un outil d'accession sociale à la propriété, et non une nouvelle forme d'investissement locatif pour les particuliers. Comprenez bien, mes chers collègues, qu'il faut absolument éviter d'entrer dans la boucle de la spéculation. C'est pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité de vendre des logements vacants à toute personne physique. J'entends déjà certains m'opposer l'argument que la possibilité pour toute autre personne physique d'acheter un logement social existe. Oui, elle existe, mais elle pose un véritable problème aucune condition n'est requise s'agissant de la situation économique et sociale de l'acheteur ; de ce fait, rien ne peut garantir que le logement continue de répondre à une vraie demande sociale, alors même que le besoin en logements est plus que primordial. Et puis, ne soyons pas dupes, nous connaissons la situation le Gouvernement veut accroître la vente de logements HLM, pour porter leur nombre à 40 000 par an. Dans le même temps, nous savons tous la difficulté actuelle à trouver des acheteurs dans le parc social. conséquent, cette situation va conduire les bailleurs à vendre les HLM aux personnes les plus aisées, qui ont la capacité financière d'investir.

permettrait donc à des promoteurs immobiliers d'acquérir des logements sociaux dont le prix de cession est librement fixé par l'organisme vendeur. Le parc de logements sociaux est constitué, en grande partie, par des financements publics. La cession de ces logements doit donc d'abord permettre l'accession à la propriété des ménages modestes et le financement de nouveaux logements sociaux par la vente à des particuliers ou à d'autres organismes de logement social, et non la réalisation d'opérations immobilières financièrement attractives pour des promoteurs immobiliers ou des investisseurs, tels que des fonds de pension. Il convient par conséquent de supprimer cette possibilité de vente à des personnes morales de droit privé.

Le projet de loi prévoit que le prix de vente des logements sociaux est fixé librement. L'avis des domaines est une garantie de transparence et de juste prix. Nous proposons donc que le prix de vente soit compatible avec l'avis des domaines, laissant une certaine marge de négociation dans le cadre de la vente.

Cela aurait pour conséquence de confier à l'Agence nationale de contrôle du logement social, l'ANCOLS, une mission de surveillance des opérations immobilières conduites par les bailleurs, ce qui n'est pas dans tels moyens humains. En revanche, un organisme de l'État se charge très bien de cette tâche depuis des décennies : le service des domaines, récemment devenu la direction de l'immobilier de l'État, de Bercy, cette dernière dispose de tous les moyens humains et de toute l'expertise nécessaires pour remplir cette mission. La DIE a toujours fait office de juge de paix objectif et constitue une référence en la matière.

Il dispose d'une méthode de calcul fiable, qui constitue une véritable référence. Quand des logements HLM sont vendus, il n'y a donc pas de raison que les domaines n'interviennent pas, c'est bien d'un patrimoine public, s'il en est, qu'il s'agit. L'évaluation des domaines garantit un prix juste et sécurise le dispositif pour l'ensemble de la chaîne. L'amendement

est, comme la République, en marche ! Je ne sais pas quel « ÉLAN » imprime à la société le présent projet de loi, mais nous avons bien l'impression que la marche sera plus difficile pour certains que pour d'autres dans les années à venir. La refonte complète de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, menée en grande partie dans l'article 29, n'aurait que des conséquences limitées, puisqu'il s'agit, dans les faits, de l'article couvrant les ventes intervenant entre organismes.

Autrement dit, moins d'un an ou presque après avoir fait de la société nationale immobilière l'opérateur de référence en matière de logement intermédiaire, le Gouvernement entend désormais suivre pour réaliser ses actifs et apporter éventuellement, sous la forme de dividendes, son concours au redressement des comptes publics. Il convient de rappeler que, à échéance de dix à quinze ce sont 800 000 logements qui pourraient être ainsi mis sur le marché, à commencer, bien évidemment, par les « meilleurs morceaux », c'est-à-dire les logements PLS et PLI, ceux dont le loyer est aujourd'hui le plus élevé et dont les caractéristiques peuvent constituer, rapidement, une source de revenus importants pour les acquéreurs, notamment pour quelques banques ou compagnies d'assurance ayant besoin de contreparties à présenter au regard de leurs engagements. On ne réglera sans doute pas la crise du logement dans notre pays avec 40 000 ventes de logements HLM par an, surtout quand il n'y en a qu'un peu moins de 10 000 aujourd'hui, mais on offrira quelques opportunités à certains. La banalisation de ces logements permettra de leur appliquer rapidement des loyers sensiblement plus élevés que ceux qui sont pratiqués dans le secteur locatif social, comme cela a été rappelé ce matin, même quand il s'agit de PLS ou de PLI, tout en faisant tomber, par exemple, le statut fiscal, ou encore le jeu des garanties appelées à l'origine. En même temps, comme l'aide à la pierre, déjà inexistante ou presque, est aujourd'hui une vue de l'esprit, il faut prévoir d'autres sources de financement de la construction sociale. Quelle place sera laissée, dans ce cadre, à la mixité sociale ?

Nous le savons, puisque nous avons exercé, pour la plupart d'entre nous, des responsabilités territoriales, les collectivités territoriales sont des acteurs extrêmement importants du logement locatif public et de la politique de l'habitat. C'est grâce à leur contribution que bon nombre d'opérations se font.

Il tend, d'une part, à porter de cinq à dix ans le délai durant lequel la personne qui a acquis un logement et qui souhaite le revendre doit en informer l'office public d'habitat ou d'HLM ayant effectué la vente dudit logement

de cet amendement me semble tout à fait logique. L'ensemble de ceux qui ont contribué à la concrétisation des opérations peut ainsi recueillir le bénéfice d'une éventuelle

de quinze ans. Cette ouverture du dispositif de vente permettra aux bailleurs sociaux de valoriser plus facilement leur patrimoine. La vente à l'unité, dans ce cas, n'intéressera pas les acteurs institutionnels privés du logement. J'ajoute que l'avis conforme

n° 765 rectifié, M. Canevet propose que l'acquéreur personne physique qui doit informer l'organisme de son souhait de revendre son logement soit tenu à cette obligation pendant dix ans, et non plus cinq ans. Si l'acquéreur personne physique réalise une plus-value de plus de 25 %, alors

enfin, à l'amendement n° 181. Je rappelle que la vente à une autre personne physique intervient bien en dernier lieu, lorsque l'on n'a trouvé ni locataire acquéreur ou personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires

Se pose la question de la gestion de ces copropriétés dont une partie des logements aura été cédée par les sociétés de vente d'HLM. La commission des affaires économiques a précisé que l'organisme HLM antérieurement propriétaire assure les fonctions de syndic, en lieu et place de la société de vente. Cette solution est bien entendu bienvenue, puisque le propriétaire dispose d'une meilleure connaissance de l'immeuble. Toutefois, il est prévu que l'organisme HLM puisse renoncer ou conclure une convention contraire. Le présent amendement a pour objet d'écarter la possibilité pour l'organisme HLM de renoncer à l'exercice des fonctions de syndic, afin d'encourager l'adoption d'une convention entre la société de vente et l'organisme HLM.

avec le nouveau partage des responsabilités dans ce domaine, notamment compte tenu des responsabilités confiées aux collectivités locales dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. Au cours des dernières années, les CRHH ont vu leur mission s'élargir

transformant progressivement cette instance de concertation resserrée autour des principaux acteurs en une assemblée au caractère plus informatif que décisionnaire. Certains acteurs se sont ainsi détournés des CRHH, devenus de simples chambres d'enregistrement pilotant à distance les directives nationales. Il conviendrait de faire évoluer les missions des CRHH autour de feuilles de route claires et de responsabilités renforcées, dans une déclinaison locale des dispositifs nationaux en faveur de l'habitat- cela fait écho aux échanges que nous avons eus précédemment. À ce titre, pour isoler la vocation consultative de CRHH largement ouverts aux différentes parties prenantes des politiques du logement d'une capacité plus rapprochée de prise de décisions concernant plus directement les acteurs locaux financeurs des politiques du logement, il est proposé de rattacher aux CRHH existants un comité des financeurs.

dimension -et, ainsi, de faciliter la mise en oeuvre de politiques du logement au plan local. Je rappelle que le souhait du Gouvernement est d'avoir, demain, des commissions régionalisées de l'ANRU

Après la présentation qui vient de nous être faite, je m'interroge cependant sur la portée de cet amendement : faut-il en déduire que la question du financement ne serait plus abordée dans le cadre du CRHH ?

Dans la pratique, les bailleurs sociaux organisés en groupes fortement « verticalisés » ou disposant d'un parc de logements répartis sur plusieurs territoires privilégient le plus souvent une logique patrimoniale. le Gouvernement s'est fixé comme objectif d'accroître la vente de logements HLM pour financer de nouveaux programmes. À cette fin est introduit un plan de vente qui sera annexé

à favoriser le développement de copropriétés dégradées, comme nous l'avons dit. Cet amendement tend à l'élaboration d'un volet territorial du plan de vente des CUS, dès lors qu'un organisme HLM est propriétaire de plus de 5 % du parc du territoire d'une collectivité. Le plan de vente des CUS ne doit pas, en effet, remettre en cause les orientations définies par le PLH. Ce volet territorial, annexe obligatoire des CUS, doit permettre de territorialiser, à l'échelle de l'intercommunalité, l'ensemble des interventions d'un bailleur social, en articulation avec le PLH. À cette fin, il comprend, pour le territoire, le programme détaillé des ventes et le plan territorialisé de prévention des risques de dégradation des ensembles immobiliers visés par le plan de vente. Il s'agit bien évidemment de disposer d'une idée très précise de ce qui constitue le volet

va dans le même sens que le précédent : il vise à assurer la cohérence entre le plan de vente des CUS et la convention de coopération annexée au programme local de l'habitat, conclue par les collectivités territoriales avec les bailleurs sociaux. Il s'agit d'ajouter des garanties, pour associer

les collectivités locales. Celles-ci contribuant activement à la production du parc social et à son évolution, il nous semble logique qu'elles soient étroitement associées au devenir du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire.

L'État doit lui aussi être associé à cette concertation et être signataire de la convention territoriale de coopération. Cette convention serait partie prenante des CUS et annexée au programme local de l'habitat.

L'objectif est d'assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l'habitat décidées par les collectivités et traduites dans leurs documents de programmation et les stratégies propres à chacun des bailleurs présents sur un territoire figurant dans leur plan stratégique de patrimoine et leur CUS.

qui comprend un volet territorial. Je rappelle, par ailleurs, que les EPCI sont signataires des CUS conclues par les organismes qui leur sont rattachés et peuvent être signataires, à leur demande, des CUS des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. Les EPCI sont également les premiers concernés par les conventions intercommunales d'attribution, s'agissant des questions de peuplement. À l'heure où l'on recherche la simplification des normes

de devenir propriétaires pour une enveloppe d'environ 800 millions d'euros. L'APL accession avait vocation à soutenir des ménages aux revenus modestes, souvent dans les zones détendues, particulièrement dans les centres-bourgs et parfois dans des zones où il n'existe pas d'offres locatives adaptées pour ces familles. Dans beaucoup de cas, le projet d'acquisition n'aurait pu être possible sans le soutien de l'APL accession qui intervenait comme un véritable déclencheur. Cette suppression n'est pas cohérente avec les objectifs du Président de la République. Pour vendre 40 000 logements sociaux à leurs locataires, il faut

quant au financement des aides à la pierre, la Fédération des entreprises publiques locales avait logiquement proposé aux parlementaires d'exclure les bailleurs sociaux des outre-mer de la part de l'assiette des cotisations alimentant ce fonds ouvert uniquement à la métropole. Néanmoins, ni le Gouvernement ni le Parlement n'ont souhaité retenir cette proposition. Face à des besoins estimés à 100 000 logements, les opérateurs sociaux sont pourtant confrontés à de multiples freins liés à la fois aux conditions et aux moyens de financement du logement, à des contraintes en matière d'offre de terrains constructibles et à des prix du logement pas toujours compatibles avec le taux d'effort des ménages modestes. Aujourd'hui, les bailleurs locaux ultramarins demandent justice fiscale en la matière : l'impact financier pour la société martiniquaise d'HLM s'élève, par exemple, à 500 000 euros par an. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet d'exonérer les bailleurs sociaux ultramarins du paiement des contributions au Fonds national des aides à la pierre, dans la mesure où ce fonds ne finance que des opérations réalisées sur le territoire de la France métropolitaine.

Le paragraphe VII de l'article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, prévoit que le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer de participer au capital de cette société à condition qu'il cède, avant le 8 août 2016, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement. Cette disposition pose une véritable difficulté en ce qu'elle ne traite pas précisément de la situation d'une entreprise publique locale exerçant plusieurs activités dont certaines continuent de relever de la compétence de la collectivité départementale.

Le présent amendement a pour objet de préciser que les départements peuvent bien évidemment continuer de détenir des parts sociales dans les SEM locales exerçant plusieurs activités et dont l'une au moins des activités inscrites dans l'objet social relève d'une des compétences que la loi lui attribue.

Nous avions voté contre ces ordonnances, considérant que la création du groupe Action Logement témoignait de la volonté de passer d'une notion de réseau à une notion de groupe. Or la richesse d'Action Logement, c'est justement son réseau. Ce dernier a largement diminué depuis 2009. Sous couvert d'efficacité, ces regroupements témoignent d'une vision plus financière que stratégique ou sociale. Il s'agit de créer le premier groupe de logements en France, fort d'un patrimoine de près de 900 000 logements.

d'en permettre la collecte à partir de dix salariés, contre vingt actuellement. Nous demandons également que l'ensemble des salariés bénéficie de ce dispositif. Enfin, les organisations syndicales demandaient, dans le cadre de la réforme, la mise en oeuvre d'un véritable paritarisme.

Ainsi, les représentants d'une des entités du groupe ne peuvent siéger dans les autres entités du groupe. Au vu du constat de manque de fluidité dans les instances et des dysfonctionnements majeurs que cela peut entraîner, cet amendement vise à supprimer les incompatibilités de cumul de mandats et de fonctions, afin de permettre aux partenaires sociaux d'Action et à la direction générale d'assumer le rôle qui leur est conféré. En outre, l'adoption de cet amendement serait l'occasion de pallier l'absence de mise en place du comité des partenaires, instance essentielle quant aux orientations et à la distribution de la PEEC, la participation des employeurs Je rappellerai le contrôle qu'a mené la commission des affaires économiques sur la réforme d'Action Logement en mai dernier. Le comité des partenaires du logement social n'a pas été installé, faute de publication des décrets relatifs à sa composition et à son fonctionnement, plus d'un an après la mise en oeuvre de la réforme. Or cette structure s'avère fondamentale dans la mesure où elle est censée jouer le rôle de vigie à l'égard des orientations et de la distribution de la participation des employeurs à l'effort de construction. par l'article 31 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, de ratifier les ordonnances prises en application de la loi du 1 juin 2016 habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer Action Logement.

donc l'objet de cet amendement, relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction a instauré des règles d'incompatibilité de mandats et de fonctions au sein des conseils d'administration entre les entités d'Action Logement. Il est apparu que les instances du groupe manquaient de fluidité et que ces règles entraînaient un certain nombre de

à ce que les textes définitifs adoptés précisent qu'une même personne physique ne pourra siéger que dans une et une seule instance. Tous les administrateurs des trois nouvelles structures seront donc distincts

amendement vise à interdire à Action Logement Groupe de « détenir ou acquérir aucun titre de capital au sens de l'article L. 212-1-A du code monétaire et financier

de portage, notamment de portage immobilier ou d'objets de construction ou de services. Action Logement Groupe est simplement

me paraît aller dans ce sens. Plus précisément, il peut le faire en son nom propre et dans sa propre activité. En revanche, il ne peut pas utiliser l'argent de la collecte pour faciliter son action de prise de participation au titre de son action de logement social,

Je propose que nous n'ouvrions pas la boîte de Pandore, pour qu'il ne vienne à l'idée de personne de requalifier le capital issu de prélèvements obligatoires

sur la contemporanéisation de la base ressource des APL. C'est un sujet et un mot compliqués, mot que nous aurons l'occasion de prononcer à de multiples reprises au cours des prochains mois.

à Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes dont l'habitat permanent est constitué d'une résidence mobile d'accéder plus facilement aux logements sociaux, en inscrivant l'accès de ces personnes à un logement bâti et adapté dans les missions générales des bailleurs sociaux. Il y va de l'intérêt non seulement des personnes sédentarisées ou en voie de sédentarisation, mais aussi des collectivités locales, qui, dans leur grande majorité, ne disposent pas des outils pertinents en termes d'habitat pour répondre à cette évolution sociétale.

code de la construction et de l'habitation, afin de favoriser l'accès à un logement bâti et adapté aux personnes dont l'habitat permanent est constitué d'une résidence mobile et qui sont en demande de sédentarisation. Je considère que le public visé

Pour mémoire, dans son rapport public annuel, la Cour des comptes relève : « le potentiel d'accueil des aires spécifiquement destinées aux gens du voyage a sensiblement augmenté, mais certaines d'entre elles accueillent des quasi sédentaires, contrairement à leur vocation qui est d'accompagner la mobilité. » Elle constate également que « l'amplification du phénomène de " l'ancrage territorial " impose de considérer le développement de l'offre d'habitat adapté comme un but de même importance importance que l'accompagnement de la mobilité. » La Cour recommande ainsi de « redéfinir les objectifs de la politique d'accueil et d'accompagnement des gens du voyage, en prenant notamment en compte le besoin d'un habitat adapté. Il y va de l'intérêt non seulement des personnes sédentarisées ou en voie de sédentarisation, mais aussi des collectivités locales, qui, dans leur grande majorité, ne disposent pas des outils pertinents en termes d'habitat pour répondre à cette évolution sociétale. Quel est l'avis de la commission ?

siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, pour présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux. La liste des organisations nationales auxquelles doivent être affiliées les associations de locataires est suffisamment large pour prendre en compte toute la diversité des familles d'associations ayant notamment pour objet la défense des intérêts des locataires. Par cet amendement, il s'agit de rétablir l'affiliation des associations de locataires à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation.

une structure à laquelle les associations indépendantes se rattacheraient. Dès lors, elles auraient la possibilité, le cas échéant, de participer aux organes de gouvernance. Cela permettrait de prendre en compte les préoccupations de chacun, en répondant

avec les objectifs du logement social fixés par le présent code », est maintenue par ailleurs. J'entends ce que vous dites, monsieur le secrétaire d'État, mais il faut entendre aussi les petites associations

Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

et un manque d'entretien des places de stationnement laissées vacantes faute de locataire. La vacance des places de stationnement est évaluée entre 25 % et 35 %. Pour remédier à cette situation sans imposer de charge excessive aux locataires fragiles, la définition d'un zonage dérogatoire pourrait être confiée au préfet. présenterait l'inconvénient d'imposer des charges locatives excessives pour les locataires en situation de fragilité financière en secteur dérogatoire. À l'inverse, en zone très dense où les places sont toutes louées, il convient de ne pas générer de pertes de recettes pour les bailleurs. Cet amendement vise donc à compléter le dispositif actuel avec un mécanisme souple fixant un montant raisonnable du loyer des aires de stationnement au-dessus duquel les locataires demeurent libres de renoncer à la location d'une aire de stationnement. Quel est l'avis de la commission ? La commission